Monsieur le président,

le 16 octobre dernier, le Sénat adoptait définitivement le projet de loi ÉLAN. C'était l'aboutissement d'un processus engagé il y a maintenant plus d'un an avec la mise en place de la conférence de consensus sur le logement, souhaitée par le Président du Sénat et acceptée par le Président de la République. l'issue de ce vote, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution des dispositions relatives, notamment, à l'accessibilité des logements et à la loi Littoral. Dans sa décision du 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, mais il a censuré d'office dix-neuf articles, parmi lesquels l'article relatif à la création d'un observatoire des diagnostics immobiliers, celui relatif aux conditions de délivrance des congés en matière de bail par une société civile immobilière familiale, celui instaurant une obligation pour le bailleur de notifier au syndic les coordonnées de son locataire ou encore celui relatif à la révision tous les cinq ans du décret fixant la liste des charges récupérables. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que ces articles n'avaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial et qu'ils étaient en conséquence contraires à l'article 45 de la Constitution. Mes chers collègues, vous le savez, le Sénat fait preuve d'une grande vigilance sur les questions de recevabilité et n'hésite pas à supprimer des dispositions introduites par l'Assemblée nationale

aucune indication dans sa décision sur le cheminement l'ayant conduit à censurer ces dispositions. Je regrette que ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'aient été consultés par le Conseil constitutionnel lors de la procédure d'examen de la saisine. Si tel avait été le cas, nous aurions sans aucun doute des arguments justifiant pleinement le lien entre ces dispositions et le projet de loi initial. La proposition de loi que je vous présente aujourd'hui tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. Je n'ai cependant pas souhaité reprendre l'ensemble des dix-neuf articles censurés. Il s'agit uniquement des articles L'article 91 a pour objet de simplifier le droit actuel en inscrivant le principe selon lequel les bailleurs sociaux accordent aux forces de l'ordre un accès permanent aux aux parties communes de leurs immeubles. L'article 121 vise à compléter le délit d'occupation des halls d'immeuble et à faciliter la résiliation du bail en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Notre rapporteur, Dominique Estrosi Sassone, vous présentera ces articles plus longuement. Naturellement, cette proposition de loi n'a pas vocation à rouvrir les débats que nous avons eus lors de l'examen du projet de loi ÉLAN. Il s'agit d'examiner deux dispositions

Reconnaissons également que cette proposition de loi ne réglera pas tous les problèmes de sécurité et de tranquillité, chacun en conviendra. Je le sais, les prises de position politiques de nos collègues seront fortes sur ce sujet. Néanmoins, il me semble important d'envoyer un signal non seulement aux bailleurs, mais aussi aux habitants de nos quartiers.

qui est l'essence même du logement social par rapport au logement privé, serait dès lors en grand danger. Comme je l'ai annoncé en juillet dernier, la commission des affaires économiques mettra en place, avec un certain nombre de collègues et de maires engagés sur ces sujets et de toutes les sensibilités politiques, un « baromètre des banlieues », qui nous permettra d'évaluer ce qui se passe réellement sur le terrain : comment nos politiques de droit commun sont-elles mises en oeuvre ? Quelles mesures correctives doivent être prises ? Pour conclure, je souhaite, monsieur le ministre, que cette proposition de loi aille au bout du processus législatif. Espérons que le Gouvernement accepte de l'inscrire rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale

qui a pour objet de reprendre le contenu des articles 91 et 121 de la loi ÉLAN, lesquels ont été censurés par le Conseil constitutionnel.

La proposition de loi comprend deux articles. L'article 1, qui reprend l'article 91 de la loi ÉLAN, pose le principe selon lequel les organismes d'HLM accordent à la police et à la gendarmerie nationales et, éventuellement, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. La commission s'est montrée favorable à cet article, qui simplifie opportunément la procédure actuelle d'autorisation d'accès des forces de l'ordre aux parties communes des immeubles du parc social. L'article 2 de la proposition de loi prévoit plusieurs modifications. Tout d'abord, le premier paragraphe vise à modifier le délit d'occupation abusive des halls d'immeuble. Il tend à sanctionner un nouveau cas d'occupation abusive des parties communes. Ainsi, l'occupation en réunion des espaces communs ou des toits des immeubles, qui nuit à la tranquillité des lieux, sera punie des mêmes peines que celles actuellement prévues pour le cas d'occupation abusive des espaces communs. En outre, la peine d'emprisonnement encourue pour le délit d'occupation abusive est aggravée et passe de six mois à un an, lorsque l'occupation est émaillée de voies de fait ou de menaces. Le juge pourra également prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction pour trois ans au plus de paraître dans certains lieux définis par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise. Il s'agit ainsi de reprendre en partie des modifications apportées au délit d'occupation des halls d'immeubles introduites dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles avaient déjà été censurées par le Conseil constitutionnel pour des motifs de forme. Le deuxième paragraphe de l'article 2 reprend des dispositions initialement introduites par le Sénat en matière de résiliation du bail du bail et modifiées par la commission mixte paritaire. Le droit actuel prévoit la possibilité d'introduire une clause permettant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Néanmoins, cette disposition ayant été introduite en 2007, les contrats de location conclus antérieurement ne la mentionnent pas, ce qui rend plus difficile l'expulsion du locataire qui ne respecte pas son obligation d'utiliser paisiblement son logement. Il est donc proposé que la clause permettant de résilier de plein droit le bail en cas de condamnation définitive du locataire pour troubles de voisinage soit réputée écrite dès la conclusion du contrat de bail. Les locataires seront ainsi traités de la même façon, quelle que soit la date de conclusion de leur bail. Le dispositif a été encadré. Ainsi, le trouble de voisinage invoqué devra non seulement avoir été constaté par une décision de justice, mais aussi avoir eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour permettre le déclenchement de la clause de résiliation du bail pour les contrats en cours. On observe de plus en plus souvent des locataires qui ne respectent pas leurs obligations, ce qui a immanquablement des répercussions sur l'ensemble de l'immeuble. Par cette proposition de loi, il s'agit d'envoyer un signal positif en direction des locataires qui respectent leurs droits et leurs devoirs et occupent paisiblement leur logement, en leur montrant que le non-respect de ses obligations par un locataire est sanctionné. L'article 2 précise en outre que sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions relatives au trafic de stupéfiants commises dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. Le contrat de bail pourra être résilié de plein droit à la demande du bailleur social, lorsque le locataire ou l'un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale aura été définitivement condamné pour l'une de ces infractions commises

estimé qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. La résiliation du bail en cas de trafic de stupéfiants va dans le bon sens. En effet, le trafic de stupéfiants est l'une des causes majeures des troubles de voisinage dans les quartiers et constitue,

passée en force de chose jugée pour résilier automatiquement le contrat de location, les bailleurs sociaux pourront engager plus facilement des actions à l'encontre des locataires qui nuisent à la tranquillité du voisinage par leurs agissements. La commission des affaires économiques a ainsi adopté sans modification les deux articles de la proposition de loi. Les nouveaux outils que nous proposons de mettre en place supposent nécessairement que toute la chaîne police-justice soit pleinement mobilisée. Lors de nos débats en commission,

En conclusion, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cette proposition de loi. La parole

Ces derniers aspirent à la sécurité et à la tranquillité, encore plus quand ils sont chez eux. Ils désirent une vie paisible où les nuisances et les violences, notamment celles qui sont liées aux trafics de drogue, ne viennent pas dégrader leur immeuble, leur cadre de vie et toute l'image des quartiers dans lesquels ils vivent.

Elle reprend le contenu des articles 91 et 121 du projet de loi ÉLAN dans la version définitivement adoptée par le Parlement. J'insiste sur ce point : ce sont des mesures que le législateur a déjà adoptées et que le Conseil constitutionnel a écartées pour des raisons

ou spécifique de la part de l'ensemble des personnes intervenant dans les procédures en question. Elles concernent également l'accès des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement aux parties communes des immeubles, pour faire des vérifications relevant de leur ressort, ainsi que l'accès des agents de l'INSEE aux boîtes aux lettres, notamment dans le cadre des recensements. La première disposition permettra d'améliorer la prévention des expulsions locatives, raison pour laquelle nous l'avions acceptée

Les offices d'HLM sont en effet en attente de mesures plus adaptées à la situation à laquelle ils sont confrontés dans certaines résidences. Il est toutefois regrettable que les copropriétés privées, notamment dégradées, ne soient pas prises en considération, car ce problème s'y pose déjà fortement, dans des conditions différentes, compte tenu

L'article 1, qui reprend l'article 91 de la loi ÉLAN, dispose que les organismes d'HLM accordent à la police nationale, à la gendarmerie, ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. Certes, l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà un cadre légal d'intervention permanente, en précisant que « les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants

et tous les ans dans les copropriétés privées dégradées. Nous soutenons cette disposition, qui participe à la préservation de la tranquillité et de la sécurité de l'ensemble des résidents et constitue enfin une réponse simplifiée et opérationnelle. L'article 2 comprend deux volets distincts. Le premier, relatif au délit d'occupation des halls d'immeuble, vise à modifier, en le complétant, le premier alinéa de l'article 121 relatif à l'occupation en réunion des parties communes nuisant à la tranquillité des lieux, à l'accès ainsi qu'à la libre circulation des personnes. à aggraver les peines encourues, qui passent de deux à six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros à 7 500 euros d'amende. Enfin, il s'agit d'instaurer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans certains lieux,

Le second volet redéfinit le champ d'application de la clause résolutoire, qui est applicable en cas de non-paiement des loyers, charges et dépôt de garantie, de non-souscription d'assurance d'habitation ou, depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, de troubles anormaux du voisinage déjà constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. En prévoyant d'étendre le champ d'application de la clause résolutoire au trafic de stupéfiants et en visant la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal intitulée « Du trafic de stupéfiants », ce texte entend prendre en considération une catégorie beaucoup plus importante d'infractions telles que l'acquisition, la détention,

que « la question de la tranquillité publique était prégnante et récurrente pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville » et souligné la nécessité, pour les services de police et de la justice, d'« amplifier leurs actions pour assurer la tranquillité des habitants dans les quartiers

Par ailleurs, cette proposition de loi prévoit expressément l'application rétroactive de la clause résolutoire pour trouble du voisinage, et notamment pour trafic de stupéfiants. Le sujet est délicat, chacun peut en convenir, et il concernera tous les bailleurs publics et privés, puisqu'il s'agit de modifier la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Observons en effet que le Conseil constitutionnel réaffirme régulièrement la protection dont doivent bénéficier les contrats légalement conclus. Celui-ci précise que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles IV et XVI de la Déclaration de 1789 ». Chaque fois qu'il a accepté une dérogation, c'était en faveur de la personne. En outre, il existe des mesures telles que les peines complémentaires, que le juge pénal peut appliquer, ou bien des mesures permettant de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour trafic de stupéfiants dans le cadre d'une procédure au fond classique. Ainsi, même si nous reconnaissons la nécessité de faire face à la situation que nous décrivent tant les bailleurs que les habitants, la rétroactivité nous paraît constituer un facteur de fragilisation du dispositif, lequel, du fait de sa nature, est déjà très sensible, en raison de son automaticité. raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression de l'alinéa 6 de l'article 2. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste et républicain partage les objectifs de cette proposition de loi, que sont notamment les indispensables droits à la sécurité, à la tranquillité publique, au libre accès, mais aussi à la libre circulation des personnes, autant d'éléments fondamentaux pour la vie quotidienne de chacune et chacun, dans le cadre des droits et devoirs pour tous. Il nous semble cependant que la dernière disposition évoquée ne peut que fragiliser le dispositif actuel. Nous voulons insister sur la nécessité d'évaluer les crédits de droit commun. comment ne pas observer que la politique de prévention est en plein délitement, alors que, nous le savons tous, il s'agit d'un élément essentiel de la politique de sécurité et de tranquillité publique ? Quel est le bilan de la police de sécurité du quotidien lancée voilà bientôt un an par le Gouvernement ? Elle devrait se déployer dans une soixantaine de quartiers de reconquête républicaine d'ici à la fin du quinquennat. Toutefois, nous l'observons d'ores et déjà, les élus sont de plus en plus sceptiques sur les gains qu'ils pourraient tirer de cette nouvelle forme de « police de proximité Ils sont aussi plus que circonspects quant à l'articulation de ce dispositif avec leurs polices municipales et craignent une recentralisation du partenariat local entre les mains des forces de l'État. Nous souhaitons donc que la grande concertation, qui devrait s'ouvrir dans les prochaines semaines sur les bases du rapport parlementaire de M. Fauvergue et de Mme Thourot, permette de renouer avec une politique de prévention, qui, depuis plus d'un an, se fait attendre. De même, nous espérons que la justice bénéficiera du déploiement de crédits de droit commun suffisants ; ceux-ci sont indispensables pour apporter les réponses rapides qui sont attendues par nos concitoyens, sachant que l'engagement, aujourd'hui- le même constat vaut pour les effectifs et les moyens alloués à la police -, n'est pas à la hauteur des besoins et des préoccupations légitimes des habitants.

là, me semble-t-il, une bonne chose, puisque nous étions, assemblées et Gouvernement, arrivés à un texte assez consensuel, qui permettait d'aller de l'avant sur un certain nombre de dossiers, dont celui-ci. La question qui se pose, pour l'essentiel, est celle de la sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens qui vivent dans ces copropriétés et dans les logements sociaux. Nous savons tous qu'il existe, malheureusement, nombre de situations absolument intolérables ; lorsque des habitants, des locataires, ne peuvent pas rentrer à leur domicile dans des conditions normales, lorsqu'ils sont confrontés- il faut le dire -à certains réseaux et comportements qui rendent au quotidien la vie dans ces immeubles difficile

collègues élus locaux se rendent compte qu'elle est indispensable. Nos forces de l'ordre, dans nos villes, dans nos quartiers,

délinquant est bien identifié, l'empêcher de revenir sur les lieux pendant plusieurs années paraît une peine complémentaire adaptée, sachant que cette

qui ont, donc, déjà été adoptés, mais qui ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, celui-ci estimant qu'ils n'avaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. Au vu de l'importance de ces dispositions, qui ont « vocation à contribuer au bien vivre ensemble et à la préservation de la tranquillité et de la sécurité des locataires », je voudrais saluer l'initiative prise par la présidente de la commission des affaires économiques en déposant cette proposition de loi, dont les objectifs sont consensuels,

Cet article prévoit en effet un accès permanent des forces de l'ordre aux parties communes des bâtiments du parc social ; il sera répondu à la demande des bailleurs sociaux, car les outils mis à leur disposition ne sont pas toujours satisfaisants pour maintenir de façon pérenne la tranquillité d'un immeuble. Ainsi, l'article 1 donne une autorisation permanente à la police nationale, à la gendarmerie et à la police municipale de pénétrer dans les halls d'immeubles détenus par les bailleurs sociaux. disposition existe déjà actuellement, mais son application est conditionnée à une demande de renouvellement des autorisations d'accès tous les six mois, ce qui, sans rendre le dispositif inopérant, le rend pour le moins complexe à mettre en oeuvre, nécessitant régulièrement une nouvelle délibération de l'office. Nous simplifions donc la procédure actuelle en posant le principe selon lequel les organismes d'HLM accordent aux forces de l'ordre une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. Des exemples, trop nombreux, ont été rappelés en commission pour évoquer l'absence de sécurité dans certains quartiers délaissés, non par manque de volonté, mais souvent par manque de moyens. Malgré la volonté des professionnels d'assurer la sécurité des populations, certaines zones de non-droit existent sur le territoire de notre République. Or cet article 1, s'il facilite évidemment la mise en oeuvre des outils existants, en permettant la présence de forces de l'ordre dans les parties communes d'immeubles,

en soirée. Néanmoins, ces dispositions ont une véritable utilité pour la préservation de la tranquillité et de la sécurité des locataires, et sont très attendues par les bailleurs.

la médiation, pour agir en amont, et de donner à la politique de prévention les moyens d'être efficace. Tous les outils qui peuvent être mis en place pour la lutte contre les incivilités et les actions en faveur de la tranquillité publique doivent s'accompagner d'une réponse judiciaire rapide. Je défends l'idée d'un équilibre entre prévention, actions éducatives et effectivité des sanctions

article 1. Les pouvoirs publics doivent donner aux services de police et de justice les moyens d'amplifier leurs efforts pour assurer la tranquillité des habitants dans les quartiers, mais les bailleurs ont également un rôle à jouer en la matière. certaines conditions doivent en effet, en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité publique, prendre des mesures permettant d'assurer le gardiennage ou la surveillance afin « d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux Les bailleurs peuvent également recourir, en complément, à des agents de prévention et de médiation, ou à des correspondants de nuit. Ces mesures, complétées par celles que nous allons voter aujourd'hui, me semblent procéder d'une dynamique collective, susceptible de proposer un cadre global, de la prévention à l'effectivité de la réponse des forces de l'ordre et de la justice.

Ainsi, l'article 2 vient compléter l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation avec un nouveau cas d'occupation abusive des parties communes d'immeubles, en incluant la nuisance à la tranquillité des lieux, et en aggravant les peines lorsque le délit d'occupation abusive est abusive est commis avec voies de fait et menaces. Par ailleurs, cet article prévoit la résiliation automatique du bail en cas de condamnation pour trafic de drogue, et l'application rétroactive d'une clause permettant de résilier le bail automatiquement en cas de condamnation pour troubles de voisinage.

de constater combien la question de la tranquillité était prégnante et récurrente pour les habitants des quartiers, partout où nous sommes passées, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest : il s'agissait vraiment d'un sujet absolument récurrent.

Si l'Assemblée nationale nous suit et adopte rapidement cette proposition de loi, ces dispositifs pourront enfin être inscrits dans la loi, après plusieurs tentatives- le Parlement avait déjà travaillé sur ce sujet et adopté des mesures quasi identiques dans le cadre de la loi relative à l'égalité et Nous abordons, je l'espère, l'acte final qui permettra la mise en oeuvre de ces mesures utiles et attendues. Le groupe Union Centriste appelle de ses voeux la mise en oeuvre effective de ces dispositions, accompagnée de la mobilisation de moyens supplémentaires et d'une vision globale susceptible de donner sens à l'ambition du « vivre ensemble, vivre en grand » ; car c'est bien par une approche globale- nous l'avons dit,

des halls de certains immeubles, affichant les prix de leur commerce sur les murs, filtrant les allées et venues, imposant leurs lois et allant jusqu'à menacer les habitants en cas de plaintes aux forces de l'ordre. Même situation à Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne : il y a quelques semaines seulement, la police de sécurité du quotidien a interpellé deux hommes pour occupation illégale de parties communes. Faute de présence régalienne, les lois de République semblent s'arrêter aux portes de certains immeubles ; elles y sont remplacées par les diktats de délinquants et de leurs économies souterraines. La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure et la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance prévoient une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende en cas de condamnation pour occupation illégale de parties communes et de halls. Cette peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende si l'infraction s'accompagne de voies de fait ou de menaces. Cependant, ces mesures se révèlent inapplicables. En l'état actuel du droit, les forces de l'ordre ne peuvent intervenir qu'après dépôt de plainte, si l'occupation entrave l'accès et la libre circulation des locataires ou empêche le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Par ailleurs, les sanctions s'appliquent uniquement en cas d'entrave manifeste à la libre circulation des personnes. Aussi sont-elles difficiles à caractériser et inapplicables.

la loi ÉLAN, renforce les sanctions en matière d'occupation des espaces communs des immeubles et autorise la résiliation du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants. Pour faciliter l'application de ces sanctions, l'article prévoit d'élargir le délit aux occupations collectives qui ont pour effet « de nuire à la tranquillité des lieux Nous avons déjà adopté ces dispositions à l'occasion de l'examen au Sénat du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Vous l'avez rappelé, madame la présidente de la commission : elles figuraient parmi les dix-neuf « cavaliers législatifs » censurés par le Conseil constitutionnel. Qu'à cela ne tienne ! Le groupe Les Indépendants soutiendrait une troisième fois cette initiative, s'il le fallait. Les zones de non-droit n'ont pas leur place au pays des droits de l'homme. Pour renforcer ce dispositif, nous défendrons un amendement visant à étendre le délit d'occupation illégale de parties communes aux occupations individuelles ayant pour effet de nuire à la tranquillité des lieux. Le droit actuel prévoit l'intervention des forces de l'ordre uniquement en cas de nuisance « de groupe »- d'où l'expression « en réunion ». Aussi des trafiquants opérant individuellement ne sont-ils pas touchés par la législation en vigueur. La criminalité organisée représente plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, selon le dernier rapport de la police judiciaire. Plus de la moitié concerne le trafic de stupéfiants. La mise en oeuvre des quartiers de reconquête républicaine et le lancement de la police de sécurité du quotidien vont contribuer, nous l'espérons, à démanteler ces réseaux et à rétablir l'ordre et la tranquillité sur l'ensemble des territoires de la République. Pour améliorer les conditions d'exercice des forces de police, nous attendons également, monsieur le ministre, la publication du décret d'application de la loi relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, promulguée le 3 août 2018. Auriez-vous des précisions à nous apporter sur la publication de ce décret ? Monsieur le ministre, nous savons que la répression ne peut être l'unique réponse à la criminalité. Pour reprendre les mots du préfet Christian Lambert, la misère est le meilleur terreau pour la délinquance ». Ces mesures répressives n'auront aucune portée à long terme si elles ne s'accompagnent pas de mesures préventives destinées à trouver des réponses à la fragmentation de notre société, à la montée des communautarismes, au décrochage scolaire et au chômage de masse. Le groupe Les Indépendants votera ce texte, mais je défendrai avec conviction mon amendement visant à rappeler que à rappeler que le critère numérique n'est pas recevable : une personne seule peut être plus agressive et violente que des personnes en réunion- j'y reviendrai.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons dans cette assemblée pour reprendre et réintroduire dans l'arsenal législatif deux articles de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, adoptée en septembre dernier. Mme la rapporteur l'a rappelé : plusieurs articles de cette loi ont été considérés par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers législatifs. Pourtant, la majorité de ces articles sont le fruit d'un consensus, sur nos travées, entre nos différents groupes, et entre les deux chambres du Parlement. Je salue donc l'initiative de notre collègue, la présidente Sophie Primas, qui a souhaité réintroduire deux dispositifs dans l'arsenal législatif ceux concernant l'occupation des halls d'immeubles sociaux et la résiliation de bail. Bien au-delà des clivages partisans, ces deux mesures répondent à l'objectif de protéger les locataires, et notamment, parmi eux, des populations fragiles. Elles répondent aussi aux attentes des bailleurs. Sur quoi portaient ces deux articles ? Le premier, qui avait été introduit par nos collègues députés, vise à permettre aux forces de l'ordre d'avoir un accès permanent aux parties communes des immeubles appartenant aux bailleurs sociaux. On mesure aisément l'intérêt de cette mesure quand on sait que certains halls d'immeubles ou parties communes de ces logements collectifs sont considérés par des bandes de jeunes, ou moins jeunes, comme leur espace exclusif, voire privatif. Nous savons- et, je crois utile de le souligner, ceci n'arrive pas que dans les grandes villes et dans les cités -que ces lieux peuvent devenir rapidement des plaques tournantes d'économie parallèle et de trafics en tout genre, où le passage des habitants de l'immeuble n'est parfois qu'à peine toléré. Nous avons pour devoir de garantir partout le respect et la tranquillité de nos concitoyens ; à ce titre, il apparaît essentiel que les détenteurs de l'autorité publique puissent accéder aisément à ces lieux sans que leur action puisse être freinée ou entachée d'illégalité.

L'article 2 de cette proposition de loi réintroduit le dispositif de l'article 121 de la loi ÉLAN et s'inscrit en parallèle de l'article 1, puisqu'il modifie le délit d'occupation des halls d'immeubles. En effet, l'occupation illicite de parties communes a pour conséquence directe de nuire à la tranquillité des lieux. Cet article aggrave les peines encourues lorsque ce délit est accompagné de voies de fait et de menaces, en le sanctionnant d'un an d'emprisonnement. Il instaure une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans certains lieux où l'infraction a été commise. Cet article comporte un deuxième volet, et ceux qui ont été maires savent que cela peut être utile : il étend à l'ensemble des contrats de location en cours l'application d'une clause permettant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice. Cette mesure avait été introduite ici même, au Sénat, en commission. Au terme de ces quelques rappels, je souhaite dire que ces mesures sont aujourd'hui essentielles dans des quartiers souvent difficiles. Elles devront être accompagnées d'autres mesures rendant possible leur application- le déploiement de la police de sécurité du quotidien doit être l'une des réponses aux problématiques que nous venons de soulever. Pour ma première discussion générale au sein de cet hémicycle, je suis ravi de vous dire que le groupe La République En Marche votera ce texte. Nous espérons qu'il sera rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin d'améliorer le bien vivre ensemble. Notre groupe soutiendra et votera également les amendements portés par nos collègues Jean-Pierre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que notre pays affronte une crise sociale liée au mal-vivre et à l'accroissement des inégalités dénoncés par le mouvement des « gilets jaunes » et par toutes celles et tous ceux qui luttent dans ce pays, le Sénat a jugé urgent d'étudier ce texte. Nous pensons que les urgences écologiques, sociales et industrielles sont autrement plus fortes, et qu'elles devraient nous emmener sur un tout autre terrain législatif pour donner de l'espoir aux quartiers populaires et à leurs habitants.

a donné naissance à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation qui est ici visé : des lois d'essence ultra-sécuritaire, contre lesquelles notre groupe s'était battu sans relâche, considérant qu'elles seraient inefficaces, car elles traitaient une conséquence sans s'attaquer aux causes. Ces lois étaient présentées comme la solution miracle contre le squat des halls d'immeubles.

Les politiques libérales ont continué de confronter les habitants de ces quartiers au chômage et au déclassement. La distension du lien social et l'assèchement des politiques publiques, notamment dans la prévention et l'éducation populaire, ont confiné la jeunesse dans de grandes difficultés, mêlant échec scolaire et défaut d'insertion professionnelle. Soyons clairs : nous trouvons inadmissible que rentrer chez soi devienne une crainte permanente et que l'occupation des halls rende la vie des habitantes et des habitants insupportable. En outre, ces faits se déroulent souvent dans un contexte qui est celui d'immeubles délabrés, de services publics supprimés ou rabotés, de commerces qui ont déserté, autant d'éléments traduisant un abandon de l'État et un recul de la République, nourrissant le désespoir des habitants et particulièrement des jeunes, qui se pensent sans avenir et sans horizon. Ceci est inacceptable et invivable pour des millions de nos concitoyens ! Quel toupet ! Mais comment ferez-vous constater ces délits, mes chers collègues, que la police ne se rend plus dans certains quartiers, car les effectifs manquent, ou que les policiers, souvent sans expérience, ont la peur au ventre en se rendant au travail ? Une question, monsieur le ministre : qu'en qu'en est-il de la police de sécurité du quotidien, annoncée à grands coups de campagne médiatique, mais que les habitants et les élus, sur le terrain,

pour assurer une chose : l'égalité républicaine. Il faut des moyens pour les politiques de prévention et de rénovation urbaine ! Il faut de véritables moyens pour la police et la justice, afin d'assurer la sécurité et de lutter efficacement contre les trafics ! Il est nécessaire de rétablir, comme nous le proposions, une police de proximité

Par ailleurs, notre législation contient déjà des dispositions pour sanctionner de telles atteintes. Il n'est pas non plus besoin d'en rajouter avec des peines de prison et des amendes doublées ! Un tel alourdissement de la sanction pénale est inadapté au public visé. La solution répressive, plus rapide et plus visible, se révèle impuissante si elle ne s'accompagne pas d'une dimension éducative. Elle risque même d'aggraver les phénomènes de délinquance. Nous estimons donc qu'il convient de renforcer et de développer des partenariats entre l'éducation nationale, les élus, les professionnels de terrain et les bailleurs sociaux. J'en viens aux clauses résolutoires au sein des baux HLM. L'état actuel du droit permet déjà aux bailleurs d'expulser les locataires pour un tel motif. À nos yeux, rendre obligatoire cette clause seulement pour le secteur HLM crée une iniquité inacceptable entre le parc social et le parc privé. Il en est de même pour la disposition permettant de rompre le bail des personnes dont les enfants auraient été condamnés pour trafic de stupéfiants. Quelle est la sanction pour les locataires du secteur privé ? Voilà encore une inégalité insupportable ! Cela rappelle la disposition législative de 2003 qui prévoyait de couper les allocations aux familles des adolescents délinquants.

d'avoir pris l'initiative de déposer cette proposition de loi, qui reprend à l'identique les articles 91 et 121 de la loi ÉLAN. Ces deux articles ont en effet été déclarés inconstitutionnels. Dans sa décision rendue le 15 novembre dernier, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions n'avaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial. C'est donc non pas le fond, mais le choix du texte support qui a été censuré par le juge constitutionnel. Les débats ayant déjà eu lieu et un consensus ayant été trouvé, il est important d'inscrire ces dispositions dans le code de la construction et de l'habitation. Ainsi, l'article 1 de la proposition de loi reprend à l'identique les dispositions de l'article 91 du projet de loi ÉLAN. Il vise à obliger les organismes HLM à accorder à la police, à la gendarmerie nationale, voire, le cas échéant,

d'accorder à la police et à la gendarmerie nationales, voire, le cas échéant, à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles. En l'état du droit, il s'agit donc d'une simple faculté, et non d'une obligation. De sorte que si les forces de police peuvent déjà intervenir, cela suppose toutefois que les bailleurs sociaux leur en aient expressément donné l'autorisation. Afin, d'une part, de préserver la tranquillité dans les immeubles d'habitation à loyer modéré et la sécurité, et, d'autre part, de simplifier le travail des bailleurs sociaux et des forces de police, l'article 1 de la proposition de loi généralise ce principe en donnant une autorisation permanente aux forces de l'ordre de pénétrer dans les parties communes. Dorénavant, il n'y aura donc plus besoin d'une autorisation des bailleurs. Les forces de police pourront intervenir et rétablir l'ordre. Adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, avec un avis favorable du Gouvernement, cette disposition a été votée sans modification par le Sénat. Simplifiant le droit existant en autorisant les forces de l'ordre à pénétrer sans avoir à solliciter au préalable les bailleurs sociaux, va assurément dans le bon sens. L'article 2 de la proposition de loi reprend à l'identique l'article 121 du projet de loi ÉLAN. Son objet est double. il modifie l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif à l'infraction d'occupation illicite en réunion des espaces communs d'immeuble. Il élargit le champ de l'infraction aux nuisances à la tranquillité des lieux et porte la peine applicable à l'infraction de voies de fait ou de menace de six mois à un an d'emprisonnement. D'autre part, il ajoute une peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les lieux dans lesquels l'infraction a été commise.

parce qu'il est extrêmement difficile de caractériser l'infraction. Sur ce point, nous espérons que la référence nouvelle aux nuisances à la tranquillité des lieux permettra de faire évoluer les choses et que le parquet saura se saisir de cette possibilité. Il faudra également réfléchir à généraliser la vidéosurveillance dans les halls des immeubles, avec transmission en temps réel des images aux forces de l'ordre, comme cela est déjà prévu à l'article L. 123-6 du code de la construction et de l'habitation. Ancien maire de Tours, j'ai pu constater que la vidéosurveillance était dissuasive et que les locataires des organismes d'habitation à loyer modéré y étaient favorables. Le bailleur social Val Touraine Habitat a ainsi conclu un protocole de coopération avec le procureur de la République, la direction de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale. Ce partenariat institutionnalisé a permis d'apporter des solutions concrètes et rapides aux troubles de voisinage. La mise en place de ce système est précédée d'une consultation auprès des habitants de l'immeuble, ce qui permet de s'assurer de leur soutien. Et les résultats sont là sont là ! L'article 121 du projet de loi ÉLAN, repris à l'article 2 de la présente proposition de loi, modifie également la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, afin de permettre aux propriétaires de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux. Comme vous le savez déjà certainement, tout acte dommageable, comme un trouble de voisinage, permet l'engagement de la responsabilité de son auteur par une action en dommages et intérêts. Une telle action en responsabilité peut également être conduite contre le propriétaire s'il est avéré que celui-ci néglige de rappeler ses obligations à son locataire. Par ailleurs, le trouble de voisinage peut également donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure pénale. Ainsi, le voisin, quel que soit son statut, d'une personne troublant la tranquillité de l'immeuble peut tout à fait légitimement intenter une action contre le fauteur de trouble ou son propriétaire peu zélé. Afin d'offrir au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a autorisé la présence dans un bail d'une clause résolutoire en cas de troubles de voisinage ayant fait l'objet d'une décision de justice. En application de cette loi, lorsque le contrat de bail comporte une telle clause, le bail peut être résolu de plein droit en cas de troubles de voisinage. Le juge n'a alors aucun pouvoir d'appréciation ; il se borne à constater l'acquisition de la clause. Introduit par la voie d'un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, la deuxième partie de l'article 121 du projet de loi ÉLAN modifiait l'article 6-1 de la loi de 1989 précitée, afin de prévoir que cette clause résolutoire de plein droit du contrat est réputée écrite dès la conclusion du contrat. Cette clause résolutoire s'appliquera donc aux contrats conclus avant l'intervention de la loi de 2007. Enfin, l'article 121 modifiait l'article 6-1, afin d'assimiler à un trouble de voisinage justifiant la résolution de plein droit du contrat de bail la condamnation passée en force de chose jugée pour trafic de stupéfiants. Il s'agit de donner la possibilité au bailleur de résilier le contrat en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants ou de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans la mesure où le bailleur est responsable civilement et pénalement du comportement de son locataire, il doit pouvoir légalement éloigner le locataire qui adopte un comportement répréhensible. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. M. Philippe

il y a parfois besoin de faire évoluer le dispositif législatif pour permettre aux forces de l'ordre d'accéder à un certain nombre de lieux dans lesquels elles ne peuvent pas entrer aujourd'hui.

un temps considérable. Au moins deux heures ! L'arrivée du tram cette année va considérablement changer la donne. Et il y aura le métro du Grand Paris.

en réunion » et d'étendre le délit d'occupation illégale des parties communes d'un immeuble à toute occupation par un groupe de personnes ou par une personne seule des espaces communs ayant pour effet de nuire à la tranquillité des lieux. Je comprends mal le critère « en réunion », que je considère comme un critère numérique au sens premier du terme. Une personne seule peut nuire à la tranquillité des lieux,

Un accès à un toit est suffisamment restreint pour qu'une seule personne puisse être un obstacle à la tranquillité des lieux. À mes yeux,

Inscrire dans la loi que la clause résolutoire est réputée écrite dès la conclusion du contrat, c'est revenir sur la protection dont doivent bénéficier les contrats légalement conclus. Et compte tenu des conséquences irréversibles de l'application d'une clause résolutoire, c'est, selon nous, encourir un risque d'inconstitutionnalité.

les relations entre bailleurs et locataires. Ces règles sont d'ordre public. Le contrat de bail s'apparente bien à une situation légale, ce qui permet d'appliquer une loi nouvelle

jusqu'à la Cour de cassation pour aboutir à une question préalable de constitutionnalité. En quoi aurons-nous rendu service au bailleur par cette rétroactivité, même si celle-ci ne s'applique pas à des faits

ne s'oppose pas à ce qu'une norme nouvelle s'applique à des situations en cours. C'est même ce que nous votons chaque année en loi de finances. Donc le contrat en cours peut être complété par une disposition légale nouvelle sans qu'il y ait rétroactivité. En revanche, ce qui serait une rétroactivité, c'est qu'une disposition pénale soit applicable à des faits commis antérieurement à son introduction. Cette rétroactivité est écartée par la rédaction du texte. L'idée

du parc HLM serait exclue de cette possibilité de sanction et qu'il faudrait environ vingt ans, compte tenu de la rotation du parc, pour que cette disposition soit applicable de façon générale. Il n'y a pas de justesse dans le raisonnement qui consiste à qualifier de rétroactivité la simple application de la loi.

J'avais également déposé, après la décision du Conseil constitutionnel, une proposition loi reprenant l'ensemble des dix-neuf articles censurés afin de préserver le travail parlementaire, objet d'un accord en Si je vous propose d'insérer ici ces trois articles, c'est qu'ils présentent tous la caractéristique de réglementer les conditions d'accès aux parties communes des immeubles d'habitation. Je ne souhaite bien évidemment pas vous inciter à l'adoption de nouveaux cavaliers. L'amendement n° 1 vise à permettre aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres particulières dans les immeubles d'habitation selon les mêmes modalités que les agents de La Poste. Il reprend la rédaction adoptée par notre assemblée sur proposition du rapporteur Marc-Philippe Daubresse et clarifiée en n° 2 vise à autoriser de manière permanente l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement. Il s'agit là d'un article inséré sur l'initiative de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann et validé en

l'intitulé de ce texte, qui deviendrait une proposition de loi relative aux conditions d'accès aux espaces communs des immeubles d'habitation. Je vous propose ainsi tout simplement de profiter de l'excellente initiative parlementaire de notre collègue pour préserver une partie de nos travaux. La

Comme le dit Mme la rapporteur, la cohérence est importante. La politique a souvent comme principale vertu de maintenir cette cohérence. Je m'associe donc à cette cohérence et j'émets un avis favorable sur ces six amendements.